avaient déjà tiré la sonnette d'alarme. Ils sont les premiers à souligner que cet individu, qualifié de « détenu particulièrement signalé », n'était pas dans la bonne prison, qu'il communiquait avec les autres détenus, que le personnel n'avait pas le temps de fouiller sa cellule et que des moyens complémentaires de sécurité, notamment des filins, étaient Forts de leur expérience, ils avaient même demandé un transfèrement urgent, demande qui n'a pas été prise en compte. Le rapport de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, dont nous avons pris connaissance ce matin, n'est pas fait pour nous rassurer. Non, cette prison, pourtant construite en 2011, prétendument moderne et sécurisée, n'était pas adaptée pour accueillir ce type de personnage ! La preuve en est qu'il est aujourd'hui en cavale. C'est d'autant plus vrai que les plans de la prison ont fuité, qu'un drone peut la survoler en toute impunité et qu'elle n'est même pas floutée sur ... Oui, je suis choquée de découvrir sur les réseaux sociaux les images filmées par un détenu, alors que les téléphones portables sont interdits en détention ! Cela laisse à penser que les échanges avec l'extérieur sont légion. Oui, je suis choquée de voir des chaînes d'information relayer cette même vidéo en faisant abstraction de toute déontologie Oui, je suis choquée de voir ce personnage dangereux incarner aux yeux de certains une sorte de héros des temps modernes et être salué sur les réseaux sociaux par une actrice écervelée, pour ne pas dire décérébrée ! Oui, je suis choquée, quand je pense à la famille de la jeune policière municipale tuée par cet homme, et en particulier à son jeune fils

cette évasion spectaculaire, qui a été préparée par un commando hors norme, a effectivement frappé les esprits ; à divers égards, on peut le comprendre. Devant une telle situation, il faut réagir avec sérieux, avec détermination, sans surenchère. Le parquet de Paris mène une enquête. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver le fugitif. En tant que garde des sceaux, je suis responsable de la sécurité dans les établissements pénitentiaires. La prison de Réau, vous l'avez rappelé, est une prison moderne. Elle a été inaugurée par le président Sarkozy en 2011. C'est une prison sécurisée. Elle est adaptée pour recevoir des détenus particulièrement signalés, des détenus particulièrement signalés, comme l'était Redoine Faïd, qui, à ce titre, relevait d'un régime de surveillance très particulier.

Dès 2018, nous avons augmenté le budget de sécurité des établissements pénitentiaires de 10 millions d'euros. Nous avons professionnalisé et renforcé le renseignement pénitentiaire ; cela est reconnu par tous. Nous avons créé des structures étanches qui vont pouvoir accueillir des détenus radicalisés. Nous mettons en place des dispositifs de brouillage des téléphones. Nous lançons un marché pour lutter contre les drones. Nous travaillons à la sécurisation des abords des établissements pénitentiaires. Le projet de loi de programmation que je vous présenterai dès l'automne traduira ces engagements pour mieux protéger les Français.

Mme la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur. L'accord auquel est parvenue l'Union européenne vendredi dernier à Bruxelles consacre un tournant dans l'approche de la gestion de l'immigration, qui relève des États souverains et demande à terme, sans doute, plus d'Europe. Ce matin, une note de Vienne, inquiétante, a été rendue publique. Si elle était confirmée, elle finirait de démontrer que nous sommes confrontés à une crise migratoire, mais aussi à une crise politique, avec la montée des partis populistes et de la droite nationaliste au sein de l'Union.

l'Europe doit accueillir des réfugiés au nom de ses valeurs, mais elle n'accepte plus une immigration clandestine incontrôlée. Aussi l'accord que j'évoquais repose-t-il sur le renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne et sur l'ouverture de centres de contrôle, où la distinction sera faite entre demandeurs d'asile et migrants économiques. Madame la ministre, le Président de la République indiquait que, n'étant pas un pays de première arrivée, la France n'avait pas vocation à ouvrir de centres de contrôle. Je vous demande donc de bien vouloir nous préciser comment la France mettra en application cet accord de principe obtenu au Conseil européen. Comment envisagez-vous l'accueil digne des réfugiés sur notre territoire et la limitation de l'immigration économique ? Les nouvelles procédures prévues dans le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie répondent-elles aux objectifs de ce nouvel accord européen ?

Cela montre la solidarité très concrète de la France avec ses voisins européens en première ligne pour les arrivées par voie maritime. M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur a d'ailleurs salué ce matin l'arrivée des 52 réfugiés débarqués du.

faute d'accord en commission mixte paritaire -, nous souhaitons faire en sorte que les situations soient examinées dans des délais raccourcis. pas d'orientation à cet égard. Dans le même temps, nous travaillons en amont avec les pays d'origine et de transit pour dissuader les départs réguliers vers l'Europe. C'est là une priorité fondamentale, d'ailleurs validée par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens.

La réponse à la situation migratoire repose sur un équilibre entre humanité et responsabilité.

un nouveau plan pour la biodiversité, visant à contrer l'appauvrissement accéléré du monde du vivant. Lors de cette présentation, vous avez rappelé la situation catastrophique provoquée par l'effondrement de la biodiversité. Je suis de ceux qui partagent votre analyse, mais nous ne pourrons véritablement avancer tant que ce constat ne sera pas très largement admis tant par les parlementaires que par vos collègues du Gouvernement.

prise de conscience précède les actes. La réunion interministérielle inédite présidée hier par le Premier ministre en témoigne : nous allons collectivement prendre notre part de responsabilité dans ce grand fléau du XXI siècle, que nous devons arrimer de manière indissociable à l'enjeu climatique.

plus de 60 % des écosystèmes s'effondrent dans le monde entier. Si nous continuons avec ce modèle de développement, qui est parfois une licence de détruire la nature, c'est 40 % ou 50 % du vivant qui aura définitivement disparu au cours du siècle. Le Gouvernement prendra

avec entrain dans l'ère de l'après-pesticides, pour tourner le dos aux sombres perspectives de printemps silencieux et aller vers des printemps joyeux et réenchantés entendre encore longtemps, longtemps les concerts d'insectes somnolents chers à Albert Camus, ainsi que « des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants », comme le disait si bien Jacques Brel ! La parole

? Cet amendement tend à remplacer les mots : « sécurité sociale » par les mots : « protection sociale ». Il porte en lui la destruction de ce grand service public solidaire et protecteur de notre population. Il porte en lui la destruction de ce système qui « vise à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail « est financé par les cotisations des employeurs et des salariés, géré paritairement par les syndicats de travailleurs et les organismes patronaux vous le savez bien, les Françaises et les Français sont très attachés à notre système de sécurité sociale, malgré les nombreuses coupes budgétaires imposées par les gouvernements successifs.

Imaginez que, l'année prochaine, à l'occasion de la réforme des retraites, nous voulions compléter le dispositif des retraites actuel par un dispositif adapté à la dépendance.

il ne s'agit nullement d'une remise en cause de la sécurité sociale. Il s'agit de faire en sorte que ce qui nous lie et nous permet d'accompagner ceux de nos concitoyens qui en ont besoin puisse être plus fort et plus durable

on peut la moderniser, la développer, mais on ne touche pas à ce qu'Ambroise Croizat qualifiait, à l'occasion de la création de la sécurité sociale, de « loi humaine et de progrès

tout était fait pour que les élus de la Nation s'en emparent, en débattent et l'amendent dans les meilleures conditions. Ce temps est désormais révolu ; permettez-nous de le regretter. En ce temps, nous examinions une loi d'envergure pendant deux, voire trois semaines.

nous plaignons non pas d'un trop-plein, mais d'un « trop mal ». Nous ne voulons pas moins travailler ; nous voulons mieux travailler, parce que nous avons le souci de faire des lois de qualité et bien écrites pour les Français : c'est l'honneur du bicamérisme. Monsieur le Premier ministre, après les dysfonctionnements du calendrier législatif de ce printemps, allez-vous établir en septembre, puis en janvier, un programme équilibré de travail et vous y tenir, pour le bon fonctionnement du Parlement, afin que le temps nécessaire au débat et à l'écriture de la loi soit respecté ? La parole est à M. le Premier ministre.

Vous indiquez finement qu'il fut un temps où tout était parfait et qu'aujourd'hui tout est sombre. C'est ce que j'ai cru comprendre de votre question, monsieur le président

Nous avons donc beaucoup de travail. Nous assumons le fait que le rythme législatif soit intense. Les débats le sont également, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

diesel a longtemps été favorisée par les pouvoirs publics, sa part dans la vente de véhicules neufs et d'occasion diminue fortement en Europe et en France. Les inconvénients du diesel d'ancienne génération pour l'environnement et la santé ont conduit les pouvoirs publics à mettre fin à une fiscalité avantageuse. Plusieurs grandes villes, comme Paris, se sont engagées à sortir du diesel. Le 15 juin dernier, le PDG de l'alliance Renault-Nissan a annoncé vouloir diviser par deux son offre de véhicules Si l'on ne peut qu'adhérer à l'objectif de préservation de l'environnement, ce « diesel » semble aujourd'hui hermétique à toute innovation, notamment à celle de l'équipementier Bosch qui permettra de réduire les émissions d'oxydes d'azote des moteurs diesel à un niveau bien inférieur à la future norme prévue pour 2020. En août 2017, les conclusions de la mission sur les conséquences industrielles et sociales du déclin des motorisations diesel étaient claires : « Bien que le diesel soit plus favorable que l'essence au regard des objectifs d'émission de CO2 et que les moteurs diesel les plus récents soient beaucoup moins polluants [ ...] la chute du diesel est inéluctable. préconisait une action volontariste des pouvoirs publics pour accompagner la reconversion des sites. En France, le diesel représente 12 000 emplois. Dans mon département, la Vienne,

les partenariats envisagés avec les constructeurs et les régions pour trouver des orientations, en termes de reconversion, permettant de préserver l'outil de travail et le savoir-faire, quasiment unique en Europe, de ces ouvriers

Les suicides, les manifestations de policiers en colère ont révélé un malaise aux causes multiples. D'où l'idée de notre collègue Gérard Longuet, relayée par notre président Bruno Retailleau, de constituer une commission d'enquête sénatoriale. Elle a travaillé cinq mois, sous la présidence de Michel Boutant, dans le consensus le plus large, sans aucun présupposé, en toute objectivité. En cinq mois d'investigations, nous avons pu constater l'étendue et la profondeur du malaise. Nous en avons aussi identifié les causes : insuffisance de moyens, locaux vétustes et même indignes, véhicules usés jusqu'à la corde, mettant en danger les personnels, équipements insuffisants. En termes

risques physiques accrus, du terrorisme aux violences quotidiennes, doublés de risques juridiques. On le voit encore à Nantes, où certains présument la bavure et commettent des violences urbaines. Policiers et gendarmes sont en quête de sens et de reconnaissance de reconnaissance, quand ils ne sont soutenus ni par leur hiérarchie ni par les magistrats ; de sens, quand ils pédalent sur un vélo sans chaîne, faute de réponse pénale adaptée. Nous proposons des solutions un rattrapage en investissement, à portée du budget de l'État ; des révolutions culturelles en termes de management dans la police, de procédure et de réponse pénales, qui ne demandent que de la volonté politique. Avez-vous, monsieur le Premier ministre, cette volonté ?

votre assemblée a rendu publiques, avant-hier, les conclusions de la commission d'enquête qu'elle a consacrée à l'état des forces de sécurité intérieure. Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, avait lui-même été entendu par cette commission d'enquête. Vous avez eu l'occasion d'analyser avec lui les causes de ce malaise.

avec 196 millions d'euros de crédits par an pendant trois ans pour la police et 100 millions d'euros pour la gendarmerie, c'est-à-dire 9 % de plus pour l'une et 5 % de plus pour l'autre. Par ailleurs, sur le plan humain, il sera créé 10 000 postes supplémentaires de policier et de gendarme au cours du quinquennat. Il va falloir conclure ! Nous avons mis en place la police de sécurité, nous avons créé trente quartiers de reconquête républicaine, nous avons renforcé les effectifs de gendarmerie.

Madame la ministre, je regrette que M. le Premier ministre ne m'ait pas répondu. Vous nous confirmez ne pas avoir pris la mesure du problème. Le problème, ce n'est pas ce que droite et gauche ont fait ou n'ont pas fait avant vous ! Vous êtes aux responsabilités, la situation est urgente et des phénomènes nouveaux

la zone économique exclusive, la ZEE, de la Nouvelle-Calédonie représente plus de 15 % de la zone économique exclusive totale de la France. Cet immense espace maritime, d'une biodiversité exceptionnelle, qui abrite la deuxième plus grande barrière de corail au monde, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est de plus en plus la proie d'actes de pêche illégale commis par des pirates venus d'Asie. Depuis mai 2016, 73 embarcations illégales ont été identifiées, 20 arraisonnées, 9 déroutées, et près de 34 tonnes d'holothuries ont été saisies. C'est à un véritable pillage des ressources halieutiques du pays que nous avons dû faire face. Pour endiguer les actions de pêche clandestine, nous disposons, en tout et pour tout, d'une frégate de surveillance, de deux patrouilleurs P400 hors d'âge et d'un bâtiment multimissions B2M.

seraient retirés du service actif en 2020. Vous avez également confirmé leur renouvellement à l'horizon 2022-2024. Je vous le dis, il serait inconcevable inconcevable de laisser l'espace maritime calédonien en proie aux pillages pendant deux ou trois ans de plus, en mettant ainsi à mal notre souveraineté. Madame la ministre, ma question est la suivante : comment comptez-vous assurer la surveillance et la protection des eaux territoriales non seulement calédoniennes, mais aussi françaises, notamment entre 2020 et 2022 ?

le Gouvernement mesure parfaitement les menaces qui pèsent sur les zones économiques exclusives d'outre-mer et, singulièrement, sur celle de la Nouvelle-Calédonie.

dix-neuf. Ce seront onze bâtiments qui auront été livrés en 2025, renouvelant en profondeur cette composante de la défense qui avait pâti des arbitrages budgétaires antérieurs. Le premier des six nouveaux patrouilleurs qui seront livrés à partir de 2022 sera déployé prioritairement en Nouvelle-Calédonie. Ce qui vous inquiète, c'est bien sûr le retrait des deux derniers patrouilleurs P400

notamment d'une frégate de surveillance, d'un bâtiment multimissions, de deux avions de surveillance maritime de type Falcon 200 et, en complément, de moyens d'observation spatiale permettant d'affiner la surveillance maritime des vastes espaces de souveraineté de la France et de cibler les interventions. Enfin, Enfin, je souligne que la France renforce sa relation avec ses partenaires du Pacifique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Nous poursuivrons et amplifierons une coopération qui permet déjà de contribuer à la surveillance de la ZEE de la Nouvelle-Calédonie.

Du 9 au 18 juillet prochains se tiendra, à l'ONU, le Forum politique de haut niveau sur le thème de la transformation vers des sociétés durables et résilientes : quarante-sept pays, dont la France, participeront à cet événement, qui rassemble société civile et politiques pour évoquer la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Notre pays est aujourd'hui moteur dans ce domaine, qu'il s'agisse de la transition énergétique et des annonces faites récemment dans le domaine des énergies renouvelables, de la préservation de la biodiversité

Au niveau mondial, de 5 millions à 13 millions de tonnes de plastique rejoignent chaque année l'environnement marin. Si rien n'est fait, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050

industriels et fédérations viennent de s'engager dans le but de tenir cet objectif essentiel en matière non seulement de développement durable, mais aussi d'emploi. Au-delà de ces premiers signataires, nombre d'acteurs sont déjà présents sur ce champ vertueux.

Cette pépite est sans conteste une illustration de cette que vous aurez à coeur, madame la secrétaire d'État, j'en suis persuadé, de mettre en avant et qui a été au centre de la restitution, ce matin, des ateliers citoyens « Votre Europe durable en 2030

le reste du monde vers le haut en matière environnementale. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Président de la République en a fait une priorité de sa politique internationale et que j'ai lancé une initiative ambitieuse

développement durable, c'est la boussole des Nations unies pour guider et accélérer les actions concrètes en faveur du développement durable dans tous les pays du monde. Si nous voulons être au rendez-vous,

aider par tous les moyens, parce que ce sont elles qui créent des emplois et qui jouent un rôle moteur pour la compétitivité de notre pays.

Ma question s'adresse à Mme la ministre des solidarités et de la santé. Madame la ministre, la facilité aurait été de vous interroger sur le report du plan Pauvreté. Mais, comme chacun ici le sait, en juillet-août, les pauvres dépensent un fric fou sur les plages Aussi ma question portera-t-elle sur ce grand malade qu'est l'hôpital public. J'ai été surpris que, en répondant au député Alain Bruneel, avant-hier, vous ayez eu des mots forts, très forts, qualifiant de « mercenaires » les médecins qui se tournent délibérément vers l'intérim et sont payés jusqu'à 2 000 euros pour Si, sur le plan éthique et moral, cette situation est des plus choquante, nous en convenons, n'en faites pas l'arbre qui cache la forêt, car elle ne saurait, à elle seule, expliquer le mal profond dont souffre notre système de santé, plus particulièrement l'hôpital public. Je n'insisterai pas non plus sur l'état de tension qui y règne, si ce n'est pour saluer l'ensemble des professionnels qui oeuvrent au quotidien, y compris à l'heure où nous parlons, et qui s'apprêtent à vivre un été dont on peut craindre qu'il ne soit celui de tous les dangers. Vous voulant rassurante, docteur, vous avez dit que l'hôpital public était « monitoré ». Quand on commence à mettre un patient sous moniteur, c'est qu'on redoute l'arrêt cardiaque ... Vous êtes loin de rassurer les acteurs de l'hôpital public, notamment celles et ceux qui auront à gérer l'afflux de patients alors même que des services seront fermés, faute de médecins. Madame la ministre, sur quels dispositifs comptez-vous vous appuyer si l'alarme du vient à se déclencher dans nos centres hospitaliers comme dans nos hôpitaux de proximité ?

de 1 milliard d'euros, afin de développer, partout où c'est nécessaire, les moyens d'apporter soins et assistance à celles et ceux qui en ont besoin. Cela n'empêche pas l'apparition de situations de tension dans un grand nombre d'hôpitaux, notamment à certains moments de l'année, en particulier l'été.

particulièrement pendant la période estivale. La ministre des solidarités et de la santé a pris la situation en main avec les agences régionales de santé. Une enquête a été réalisée fin mai

Les Républicains. Ma question s'adressait à M. le Premier ministre. Voilà quelques jours, le Président de la République a présenté les contours du service national universel. En mars 2017, le candidat Emmanuel Macron annonçait que le service national universel serait encadré par les armées et la gendarmerie nationale, afin de pouvoir disposer d'un réservoir complémentaire de la garde nationale. Aujourd'hui, nous apprenons que ce dispositif n'a plus grand-chose de militaire. Le candidat Emmanuel Macron annonçait une durée de service comprise entre trois et six mois. On parle désormais de deux stages de quinze jours ... Je commence à douter du fait que ce service sera vraiment national et vraiment universel. Alors oui, il y a des points positifs

La cohésion nationale est une valeur que l'on ne peut pas inculquer à notre jeunesse en l'espace d'un mois. Si ce projet de service national universel devait en rester là, alors il vaudrait mieux l'abandonner et renforcer les dispositifs existants, tels que le service civique, la préparation militaire découverte et la préparation militaire supérieure. On ne peut pas imaginer dépenser plus de 1,5 milliard d'euros par an pour un outil dont la portée et l'utilité en termes de sécurité nationale seront plus que limitées. Monsieur le Premier ministre, madame la secrétaire d'État, le Gouvernement entend-il revoir sa copie concernant le service national universel, afin de créer un dispositif efficient et adapté aux réalités de la France de 2018 ?

vous posez une question difficile. Vous avez parlé des engagements du candidat Emmanuel Macron, mais je crois me souvenir que tous les candidats s'étaient engagés sur un tel projet, sans qu'aucun décrive, d'ailleurs, ce qu'il souhaitait faire ni quels moyens il y consacrerait.

Dans le cadre de la loi de programmation militaire, le Sénat a voté des crédits supplémentaires pour permettre la mise en place du service national universel. Je tenais à le rappeler.

Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. Notre collègue Michèle Vullien l'a souligné avant moi, le détenu qui aurait dû être le plus surveillé de France s'est de nouveau fait la belle, dans des circonstances consternantes pour notre système pénitentiaire et, par là même, pour votre ministère. Cette prison modèle n'en était pas une,

Le personnel pénitentiaire a été ainsi mis en situation de grand danger. Depuis dimanche, vos déclarations, plutôt convenues, ne sont pas rassurantes. La réponse que vous avez faite tout à l'heure ne l'est pas davantage. Avez-vous réellement besoin d'une enquête de quinze jours pour comprendre ce qui s'est passé et, surtout, pour réagir ? Des images tournées par des détenus et circulant sur internet nous renseignent déjà sur le déroulé de cette évasion à la James Bond ... Comment comptez-vous, madame la ministre, faire évoluer le système pénitentiaire et toute la chaîne pénale après cet événement d'une gravité exceptionnelle ? Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur Lefèvre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je tirerai toutes les conséquences du rapport d'inspection qui me sera présenté.

pour engager des politiques en faveur de la sécurité de ces établissements, qui sont destinées à prévenir ces évasions. La direction de l'administration pénitentiaire, à ma demande, travaille selon trois axes

en place des systèmes d'affectation des détenus dans des établissements correspondant à leur profil- c'est tout le travail de construction d'établissements pénitentiaires adaptés que nous effectuons enfin, accomplir des efforts importants pour la sécurité des établissements. Et je vous cite là seulement quelques actions que nous entreprenons. Nous privilégions la vidéoprotection, les dispositifs anti-projection, les dispositifs de détection, notamment de métaux, la sécurité aux abords des établissements, les équipements de sécurité pour les agents. Nous travaillons Nous travaillons également pour lutter contre le fléau des téléphones portables : nous avons passé un nouveau marché de brouillage des téléphones pour éviter les communications illicites. Son déploiement est en cours et se poursuivra à l'automne. Toutes ces mesures, qui nécessitent des moyens importants, seront confirmées par la loi de programmation que je vous présenterai. Elles s'accompagnent en outre d'un important effort en termes de recrutement de personnels. Nous nous engageons sur

n'est pas assurée, qui va se porter candidat ? Plus que jamais, les revendications des organisations syndicales du début d'année sont d'actualité. De nouveau, je veux vous interpeller sur la prolifération des portables en prison. Plus de 20 000 ont déjà été saisis depuis le mois de janvier. À Fleury-Mérogis, cinquante-six téléphones et objets connectés ont été trouvés dans une même cellule : une vraie téléboutique

La population carcérale a évolué ; elle est plus violente, plus jeune, pour partie radicalisée et désormais toujours connectée. Madame la garde des sceaux, il est urgent de proposer dans ce domaine des solutions vraiment efficaces et pérennes. La parole est à M. Jean-François Husson, pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Comme beaucoup, j'ai la conviction qu'il n'y a pas d'économie forte sans industrie forte. Or l'industrie française n'occupe pas la place qui devrait être celle de la cinquième puissance mondiale. Le déficit commercial de notre industrie s'accroît et nuit à la compétitivité économique et à l'emploi. La politique industrielle de la France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle est trop souvent abordée pour dénoncer ses insuffisances lorsque les projecteurs médiatiques sont braqués sur des dossiers brûlants : Alstom à Belfort, Arcelor Mittal à Florange, les Conti, sans oublier Whirlpool à Amiens et bien d'autres. Votre gouvernement a, dans ce contexte, une responsabilité importante, Il doit afficher une politique industrielle ambitieuse, toute entière tournée vers la modernisation de notre industrie, s'inscrivant dans les objectifs de transformation et de transition écologique que vous affichez. Dans mon département, au sein de l'espace métropolitain du Grand Nancy, la vallée du sel compte 5 000 emplois industriels, directs et indirects. Le Gouvernement a lancé en août 2017 un appel d'offres biomasse, auquel la société Novacarb, forte de 1 300 emplois, a répondu. Il vise à substituer la biomasse au charbon comme énergie pour assurer la pérennité et le développement d'une unité de production de bicarbonate plus que centenaire, avec, à la clé, la création de 100 emplois. Or la réponse se fait toujours attendre, malgré une mobilisation générale unanime en faveur de ce projet.

je vous rejoins volontiers lorsque vous dites qu'il est difficile d'envisager l'avenir d'un pays comme la France, sa force et sa puissance, sans une industrie compétitive. Je le crois profondément.

par elles-mêmes- nous considérons en effet que la logique des filières industrielles est probablement la plus féconde pour développer la compétitivité de notre industrie -, de simplification des normes applicables,

les produits de cession de certaines participations de l'État au capital de grandes entreprises -et de réduction de la fiscalité applicable au monde de la production en général et à l'industrie en particulier, avec notamment une perspective de diminution de ce que l'on appelle la fiscalité de production.

Le cas que vous évoquez, celui de la vallée du sel et de l'appel d'offres qui a été lancé, s'inscrit dans un certain nombre de programmes envisagés par les gouvernements successifs, dont l'idée est de faire en sorte que nous puissions

l'appel d'offres conduirait à un engagement d'environ 850 millions d'euros d'argent public, pour une solution qui créerait une centaine d'emplois.

comme ils doivent l'être, et effectivement employés pour servir la compétitivité de l'industrie française. En vérité, monsieur le sénateur, je n'en suis pas sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au préfet

avec l'entreprise et les autorités publiques locales pour trouver des solutions efficaces, peut-être moins triviales que cet appel d'offres, pour soutenir cette entreprise et préserver le développement industriel français. La parole est à M.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue André Pourny, qui fut sénateur de la Saône-et-Loire de 1986 à 2004.

Acte vous est donné de ces mises au point, mes chers collègues. Elles seront publiées au et figureront dans l'analyse politique des scrutins. Nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

pour prendre en compte les « raids numériques », c'est-à-dire la publication par plusieurs auteurs différents de propos sexistes et violents proférés une seule fois à l'encontre d'une même cible. Des faits récents visant des journalistes ont montré que les « raids numériques » et, plus généralement, le cyberharcèlement sont un réel enjeu de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces agressions ne sont en rien virtuelles et sont tout aussi graves que des violences physiques. Elles présentent par ailleurs des spécificités qui les rendent encore plus nuisibles pour les victimes, notamment la difficulté à identifier des agresseurs protégés par leur anonymat et le potentiel de diffusion élargi des contenus. Or la définition actuelle du harcèlement, qui suppose la répétition, ne permet pas de réprimer de tels agissements, puisque les auteurs des « raids » réitèrent rarement les mêmes propos, mais se coordonnent afin de cibler, de manière collective, la même personne. Il était donc important de combler ce vide juridique, pour sanctionner des agissements qui peuvent se révéler d'une violence extrême. Dans le même esprit, l'article 3 crée une circonstance aggravante lorsque le harcèlement sexuel est commis par le biais d'un moyen de communication électronique. Enfin, la commission des lois a introduit à l'article 3 une disposition conférant de nouvelles obligations aux plateformes et aux hébergeurs sur internet, afin de mieux lutter contre le cyberharcèlement.

environnemental ou d'ambiance. Sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes et vulgaires qui lui deviennent insupportables. Ce n'est pas du harcèlement sexuel, mais du harcèlement d'ambiance sexiste. L'Assemblée nationale

n° 114 rectifié. L'article 3 du présent projet de loi visait à renforcer la définition du harcèlement. Le texte transmis par l'Assemblée nationale comportait les mots « sexuelles et sexistes La commission des lois du Sénat a préféré supprimer le terme « sexiste », estimant que seul le harcèlement sexuel méritait de figurer dans la loi. Les membres du groupe CRCE s'opposent bien évidemment à cette logique, qui nie la souffrance des femmes au quotidien. Les violences faites aux femmes ne sont pas seulement physiques, elles passent aussi par ces comportements machistes banalisés, ces remarques blessantes et humiliantes qui visent à rabaisser les femmes, car elles sont femmes.

qui donnerait plutôt envie de pleurer. Le harcèlement doit être aujourd'hui défini le plus précisément possible dans notre droit. Ainsi, la loi ne saurait ignorer ces brimades journalières que sont les remarques sexistes, qui participent au sentiment de honte qu'éprouvent de nombreuses femmes. Cette honte, mes chers collègues, doit impérativement changer de camp ; elle ne doit surtout plus être l'apanage des femmes qui aspirent simplement à vivre dans une société égalitaire et paritaire avec leurs concitoyens masculins. Le présent amendement vise donc à rétablir dans son état initial le présent article en mentionnant expressément le caractère sexiste que peut revêtir le harcèlement. La pour présenter l'amendement n° 132. Je ne reviens pas sur la démonstration qui a été faite : je rejoins tout ce qui vient d'être dit par les sénatrices Esther Benbassa et Laurence Rossignol. J'ajoute qu'un harcèlement peut être sexiste sans être sexuel. Il est donc important pour nous de rétablir les mots « ou sexistes » dans la définition du harcèlement sexuel, afin d'harmoniser cette rédaction

les propos sexuels et les propos sexistes, qui regroupent des réalités différentes. Ils sont d'ailleurs sanctionnés sur la base d'infractions différentes. Avec ce projet de loi, nous faisons une réelle différence entre les faits de harcèlement sexuel Ces derniers doivent être réprimés par le délit d'outrage sexiste, qui répond à la même définition que le harcèlement sexuel, mais sans l'exigence de répétition, et qui concerne les propos à caractère sexiste. En effet, comme l'ont souligné le Défenseur des droits, des magistrats et des universitaires que nous avons entendus, cette extension du harcèlement sexuel aux faits sexistes entraîne une confusion entre le harcèlement sexuel et l'outrage sexiste, créé par l'article 4 du projet de loi, alors que la notion de harcèlement sexuel doit rester clairement distinguée des autres infractions. De plus, l'absence de clarté entre les deux définitions pourrait créer un risque de déqualification du délit de

hémicycle. Vous voulez absolument que l'outrage soit sexiste et que le harcèlement soit sexuel, mais il y a aussi un harcèlement sexiste. Cette misogynie au quotidien mérite

en effet que la lutte contre les propos haineux sur internet et la régulation des contenus illicites relève d'un autre vecteur législatif, qui serait plus approprié. Nous croyons qu'il incombe aux hébergeurs et aux réseaux sociaux de prendre leurs responsabilités. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux

de la commission ? Cet amendement vise à inclure une obligation de sensibilisation au cyberharcèlement dans le cadre de la formation d'initiation à la technologie et aux usages numériques. Nous sommes favorables à cette précision très utile. La commission

Cet article est l'une des mesures phares du gouvernement, à savoir la création d'une nouvelle infraction d'outrage sexiste, conçue pour lutter contre le harcèlement de rue et surtout pour le sanctionner. La commission des lois du Sénat a modifié cet article. Elle a notamment transformé la contravention prévue en un délit puni d'une amende de 3 750 euros. Pour ma part, même si je suis assez dubitative, comme l'ensemble des membres de mon groupe, sur la mise en place effective de cette infraction du fait de la nécessité nécessité de flagrance et surtout du manque de moyens accordés aujourd'hui aux officiers de police, je suis convaincue, en revanche, que pour être efficace cette infraction doit être élargie en délit autonome d'agissement sexiste. Là aussi, un interdit doit être plus clairement indiqué à la société, pour que de tels comportements et de tels propos à l'encontre des femmes cessent. Bien évidemment, au-delà de la sanction, je reste persuadée que la prévention et l'éducation à la sexualité et à l'égalité filles-garçons sont plus que fondamentales. Ce combat mérite d'être mené,

ou dépositaires de l'autorité publique. Cette qualification s'inspire de l'agissement sexiste, défini par l'article L. 1142-2-1 L. 1142-2-1 du code du travail et par l'article 6 de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, de sorte que ce délit est défini à la fois par le droit du travail et le code pénal, de même que le harcèlement sexuel est traité à la fois par le code pénal et le code du travail. La parole

que proposent les auteurs de ces amendements identiques, il n'apparaît pas souhaitable d'étendre le champ d'application du délit d'outrage sexiste au-delà de la sphère publique. Imagine-t-on sanctionner d'une peine délictuelle de simples propos outrageants tenus à titre privé ? Je rappelle que l'injure sexiste existe déjà. L'outrage sexiste doit se différencier de ce délit. Concernant les faits commis au travail,

prévues par l'article 433-5 du code pénal, il n'apparaît pas pertinent et poserait un problème d'intelligibilité de la loi pénale. Il n'est pas possible de renvoyer à des peines différentes pour un délit constitué de faits différents, même si les deux délits se dénomment « outrage ». En effet, ils n'ont en commun aucun élément constitutif de l'infraction. soit le délit poursuivi est un délit d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et les peines encourues sont prévues à l'article 433-5 du code pénal, soit le délit poursuivi est un délit d'outrage sexiste, et les peines encourues sont celles prévues par le projet de loi. Le procureur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

toute situation jugée de nature à créer un climat humiliant, offensant, dégradant pour les femmes. De toute évidence, de mon point de vue, refuser de serrer la main d'une femme crée ce caractère humiliant et dégradant, comme vous l'avez parfaitement relevé. À cet égard, nous considérons que cette partie de votre amendement est déjà

que le problème soulevé par notre collègue est bien réel. À partir du moment où son amendement est étroitement circonscrit à son objet même, je pense que nous devrions l'adopter.

-, des hommes refusaient de serrer la main des femmes, pour des raisons qui leur appartenaient, qui sont forcément respectables, et que cela induisait dans les rapports de travail une atmosphère

pour le, pardonnez-moi cet anglicisme, de l'entreprise elle-même. Je crois que nous rendrions un grand service aux employeurs en posant que ces attitudes à l'évidence sexistes entrent

qu'est-ce qu'un comportement imposé qui crée une situation intimidante, hostile ou offensante ? L'auteur de l'amendement peut-il m'éclairer

que c'est effectivement un outrage sexiste que de refuser de serrer la main des femmes par principe. En revanche, il y a des gens qui ne veulent pas serrer la main d'une femme en particulier, ou d'un homme en particulier, parce qu'existent entre eux des malentendus. Il y a une différence qui est parfois difficile à cerner.

qu'il s'agisse de l'agissement sexiste, tel qu'il est défini dans le code du travail, ou de l'outrage sexiste, tel que nous en proposons une définition dans ce projet de loi, il faut se demander si cette femme est traitée différemment

qui, ensuite, ne serviront strictement à rien. On se sera peut-être fait plaisir quelques instants, mais Mme Borne, si elle est un jour de nouveau directrice de la SNCF, pourra revenir voir le président de la commission des lois, qui n'aura toujours pas de bonne réponse à lui donner.

Ce dispositif, issu de la loi Rebsamen de 2015, ne se trouve pas dans les parties du code du travail relatives aux harcèlements et aux discriminations, mais dans la partie relative aux inégalités professionnelles.

L'article 132-20 du code pénal dispose que les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l'exception des amendes forfaitaires, peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration est destinée à financer l'aide aux victimes. Cet amendement, porté par la Fondation des Femmes, a pour objet de proposer que cette « sur-amende », en matière de sanction pénalisant des violences sexuelles ou sexistes, aide à financer la lutte contre ces comportements, et ce par l'intermédiaire des associations qui luttent quotidiennement contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. L'idée est qu'en complément des subventions de l'État et des collectivités territoriales, c'est-à-dire de la solidarité nationale, les auteurs d'infractions condamnés puissent contribuer pécuniairement au financement des services gratuits dont bénéficient les personnes victimes, comme l'accompagnement par les associations à tous les stades de l'enquête, ce qui est possible depuis La majoration des amendes affectée à l'aide aux victimes relève d'un système cohérent de contribution des auteurs d'infractions à l'aide aux victimes. de la commission ? Cet amendement vise à préciser que le montant des sur-amendes, actuellement destiné à financer l'aide aux victimes, pourrait également financer la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes. Cette disposition est avant tout cosmétique, puisque c'est une indication du

En l'occurrence, vous proposez de préciser que cette majoration financerait la lutte contre les violences sexuelles ou sexiste à travers le financement d'un certain nombre d'associations. Nous pensons qu'il n'y a pas de raison de mentionner dans cet article général, qui s'applique à toutes les condamnations, quelle que soit la nature de l'infraction, tel ou tel

des magistrates et des magistrats, des avocates et des avocats, qui nous ont indiqué se trouver parfois démunis, en matière de textes de loi, pour pouvoir sanctionner comme il se doit un phénomène appelé

croissant, notamment dans les transports en commun. L'objet de cet amendement est de combler une lacune de notre droit pénal, qui a été relevée par les nombreux praticiens que j'évoquais, en permettant de réprimer les personnes qui, notamment dans les transports, utilisent leur téléphone portable ou de petites caméras pour filmer l'entrejambe de femmes, lorsque celles-ci sont assises ou debout, et en jupe. Juridiquement, la qualification de ces faits est problématique, puisqu'il ne peut s'agir d'agressions sexuelles. En effet, il n'y a pas de contact direct entre l'auteur et la victime. Il n'y a pas non plus d'atteinte à la vie privée par captation d'images présentant un caractère sexuel, les faits se déroulant dans l'espace public. C'est ce qui est objecté, en général, lorsqu'il y a judiciarisation de tels agissements. Par défaut, actuellement, dans la majorité des cas, ces faits sont poursuivis sous la qualification de violences. Toutefois, en droit, la violence suppose,, un choc, et si la victime ne s'aperçoit de rien, le choc, même émotif, ne peut être caractérisé en droit. Nous pensons qu'il convient de réprimer ces faits, qui peuvent également survenir lors d'essais

aggravantes. Notre objectif, avec ce projet de loi, est de mieux condamner le spectre ou le continuum des violences sexistes et sexuelles et de combler les lacunes du droit relatives à des violences sexistes ou sexuelles, notamment en

? En fait, il aurait été préférable de viser chaque infraction individuellement et d'en faire une circonstance aggravante, comme lorsque les faits sont commis sur un conjoint.

Les mutilations génitales féminines, dont l'excision est la forme la plus connue, portent gravement atteinte à l'intégrité physique et psychosexuelle des femmes, des adolescentes et des fillettes qui en sont victimes. Elles constituent une violation fondamentale de leurs droits, tels qu'ils sont énoncés dans de nombreuses conventions internationales, notamment dans la Convention relative aux droits de l'enfant et dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cet amendement vise à préciser de manière explicite dans le code pénal que les mutilations sexuelles féminines, commises en France ou à l'étranger, par des résidents sur le territoire national, seront punies de dix ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende, et jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la mutilation est commise sur un mineur de quinze

L'ajout de cette précision visant à inclure notamment les mutilations sexuelles féminines ne paraît pas utile. Il pourrait même être contre-productif, ouvrant une longue liste d'exemples qui ne serait jamais exhaustive.

Considérant par ailleurs le très fort tabou qui plane sur les actes de pédophilie, ils veulent contribuer à le briser, en particulier auprès des professionnels qui interviennent dans les services des conseils départementaux en charge de l'aide sociale à l'enfance. Quel est l'avis de la commission

de femmes, dont 44 millions de moins de quinze ans. Mes chers collègues, la France n'est pas épargnée. Nous avons entendu tout à l'heure les chiffres qui ont été donnés : jusqu'à 60 000 victimes en France, même si notre pays a

pour lutter contre ces violences et les prévenir, de renforcer la vigilance par une formation spécifique de tous les professionnels en contact avec ces jeunes filles,

en précisant les missions des services de l'aide à l'enfance dans le code de l'action sociale et des familles. Plus largement, madame la secrétaire d'État, nous souhaitons vous alerter sur l'urgente nécessité de constituer une structure interministérielle qui sensibilise l'ensemble de nos institutions, afin de mener une politique conjointe coordonnée de prévention et de lutte contre la pédophilie auprès des prescripteurs institutionnels, des services régaliens de l'État et de toute autre organisation en lien avec les enfants. Les abus sexuels commis par des personnes ayant un lien d'autorité sur les mineurs traumatisent les victimes, causant des dommages psychologiques à long terme, pouvant les conduire à se mettre en danger par des conduites addictives, dépressives, voire les pousser au suicide. Cette souffrance est accentuée par le déni de justice qui résulte du fait que, le plus souvent, la loi du silence des institutions et employeurs protège, de fait, l'agresseur au détriment de la victime. Ces barrières institutionnelles s'ajoutent aux réticences des victimes à voir

pédocriminalité. Ces lignes directrices relèvent plutôt du Gouvernement, de la Direction générale à la cohésion sociale, et non du service social à l'enfance de chaque département. Cette réponse technique conduit la commission à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

la commission ? Je comprends l'intention des auteurs de ces amendements. Néanmoins, il semble un peu disproportionné de dissoudre des associations qui propagent des idées ou des théories tendant à justifier la discrimination entre les sexes. En effet, nombre de religions ont parfois des théories pouvant inciter à la discrimination en raison du sexe d'une personne. Faudrait-il pour autant interdire ou dissoudre de tels groupements ou associations ? Cela me semble une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, notamment des opinions religieuses. Je rappelle que les propos, et non pas les théories, qui appellent explicitement à la discrimination en raison du sexe de la personne

Le scrutin est ouvert.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

une telle disposition irait à l'encontre de la volonté d'avoir une sanction rapide et effective. Elle empêcherait le recours à des modes simplifiés de poursuite ou de jugement. On ne peut pas vouloir à la fois la verbalisation en flagrant délit et la constitution de partie civile Toutes les personnes entendues, que ce soit les magistrats ou les policiers, ont dénoncé une usine à gaz, quand il s'agissait d'autoriser la constitution de partie civile d'associations pour juger une contravention. Par conséquent, la commission émet

Ce projet de loi comporte de nouvelles sanctions pénales, mais aucun volet préventif, alors même que vous-même, madame la secrétaire d'État, déclariez en février dernier que si la loi « a pour but de sanctionner les violences sexistes et sexuelles, cela ne va évidemment pas sans prévention, sans pédagogie et sans communication ». La prévention des violences et de l'éducation à l'égalité et à la sexualité est une préoccupation récurrente de la délégation, comme en témoignent ses nombreux travaux sur ce sujet.

Cet amendement vise donc à renforcer la prévention des violences faites aux femmes en rendant effectives les trois séances d'éducation à la sexualité prévues par l'article L. 312-16 du code de l'éducation et en intégrant à ce dispositif une information consacrée à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour ce faire, je vous propose une réorganisation de la section 9 du titre I du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, en préservant tous les modules d'enseignement existants et en renforçant la cohérence de leur cadre légal.

la question de la sexualité est plus délicate à aborder auprès de jeunes tourmentés par les difficultés de l'adolescence. Ainsi, comme l'a relevé le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et inégalement mise en oeuvre. Ces séances d'éducation à la sexualité sont globalement insuffisantes et inadaptées. Selon l'enquête du Défenseur des droits menée auprès de 3 000 établissements scolaires, publics et privés, quelque 25 % des écoles répondantes, contre 4 % des collèges et 11,3 des lycées, déclaraient n'avoir mis en place aucune action ou séance en 2014 et 2015. Le Défenseur des droits plaidait dans son dernier rapport d'activité pour la mise en oeuvre obligatoire de ces séances

Les lacunes sont également grandes en matière d'égalité des sexualités, de respect des orientations sexuelles et des identités de genre et de lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes. L'éducation à la sexualité constitue un levier de lutte contre les discriminations et ne doit pas être réduite aux dimensions physiques et biologiques. Elle doit être appréhendée de manière globale et doit contribuer,

vote. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je souhaite réagir à l'intervention de mon excellente collègue Annick Billon. Je partage en général ses points de vue, mais je trouve qu'elle oublie là un partenaire essentiel : entre l'éducation nationale et la pornographie numérique, il y a les parents,

Pour être agréable à ceux qui prennent le train, je serai très brève. Le présent amendement a pour objet d'élargir les possibilités de délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes victimes de violences exercées dans l'espace public, sur leur lieu de travail ou au sein de la famille, lorsque la personne est partie prenante à une procédure civile ou pénale liée aux violences.

ou à l'étranger menacé de mariage forcé ou de mutilations sexuelles, ainsi qu'aux personnes victimes de traite des êtres humains. Cette question a déjà été débattue lors de l'examen du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, au cours duquel la commission des lois du Sénat a défendu les droits des femmes. De plus, cet amendement est satisfait par les dispositions actuelles relevant du droit des étrangers, qui prévoient déjà la délivrance de titres de séjour aux femmes victimes de violences conjugales ou encore aux étrangers victimes de traite des êtres humains. du droit d'asile, le CESEDA, envisage la délivrance et le renouvellement des cartes de séjour des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales. L'article L. 316-1 du même code prévoit qu'est délivrée à l'étranger victime de traite des êtres humains, qui porte plainte ou témoigne, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». prévoit également la délivrance d'un titre de séjour temporaire à l'étranger bénéficiaire d'une ordonnance de protection en raison de violences exercées au sein du couple. Le CESEDA est même plus protecteur que l'amendement proposé, car il prévoit la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles après un certain délai. En outre, je rappelle que les violences commises dans l'espace public

Cet amendement vise à reconnaître le statut de réfugié aux femmes persécutées ou menacées de persécutions dans leur pays, en raison de leur action en faveur des droits des femmes, du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes,

mais nous ne sommes pas totalement satisfaits du champ de protection, trop restreint à nos yeux.

octroie déjà l'asile à « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. » Sont ensuite énumérés les différents éléments constitutifs de la politique de santé, comme la préparation et la réponse aux alertes et aux crises sanitaires, ou encore la prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d'autonomie. Nous proposons que soit expressément inscrit dans la loi que la prévention des violences faites aux femmes fait partie intégrante de la politique de santé publique menée par l'État. Les violences conjugales continuent de tuer dans notre pays. Ainsi, au moins 109 femmes en sont mortes en 2017, et ce chiffre ne tient pas compte des suicides consécutifs à des violences ou à des menaces. L'enjeu de santé publique, pour toutes ces femmes, ne fait pour nous aucun doute. Il vaut mieux repérer et mettre en sécurité les femmes victimes de violences conjugales. Il faut permettre une utilisation plus importante du dispositif « Téléphone grave danger ». Il faut encore renforcer les moyens des associations, développer les lieux d'hébergement les lignes d'écoute. Ce qu'il faut, finalement, c'est une politique ambitieuse sur tous les aspects de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et surtout une politique qui se donne les moyens de ses ambitions. Quel

Les gouvernements successifs ont présenté des plans de lutte contre les violences faites aux femmes et un plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Le rôle du Parlement est de suivre

Mes chers collègues, je vous le dis, comme toujours je l'espère, avec beaucoup de respect et de courtoisie : la loi organique relative aux lois de finances renvoie à la loi le soin de déterminer la liste des annexes obligatoirement jointes chaque année au projet de loi de finances initial,

du Gouvernement ? Je partage évidemment la volonté d'évaluer ce qui est fait et de rendre compte des avancées des différents plans. C'est pour cette raison que, à partir de la rentrée

du cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes et du premier plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Vous nous avez répondu que ce suivi était bien entendu déjà prévu dans le cadre de l'évaluation des engagements du Président de la République. Je souhaite naturellement que les engagements du Président de la République soient tenus et évalués, mais pourriez-vous me confirmer

d'excellente qualité, me semble-t-il, puisque nous avons su, dans une atmosphère très respectueuse des uns des autres, échanger sur des sujets difficiles et rechercher les meilleurs voies et moyens pour atteindre l'objectif que nous partageons tous. Le projet de loi, dont nous attendions beaucoup, nous a déçus d'emblée.

au report du délai de prescription à la majorité de la victime, à l'amélioration des notions de violence, de menace et de surprise, au droit à l'enregistrement audiovisuel pour toutes les victimes, au renforcement de l'obligation de signalement de mauvais traitements sur mineurs,

L'intensité et la qualité des débats de ces derniers jours reflètent l'implication de chacun à mieux protéger les mineurs victimes de violences sexuelles. Il est vrai que nous ne nous accordons pas sur les moyens à mettre en oeuvre pour y participer. Je souhaite néanmoins saluer un texte porteur d'avancées majeures, à l'instar de l'allongement du délai de prescription de vingt à trente ans, de la répression du harcèlement de rue, ainsi que de la condamnation des « raids numériques ». Je me félicite tout particulièrement que notre chambre ait pu amener le Gouvernement à revoir sa position sur la notion d'atteinte sexuelle avec pénétration. Il s'agit d'une décision importante, qui fait écho aux doléances de nombreux experts, pour la protection des mineurs. Je me réjouis par ailleurs que l'amendement de notre collègue Laure Darcos visant à renforcer la protection des personnes particulièrement vulnérables, comme les sans domicile fixe, ait été adopté. C'est l'un des amendements émanant de

hostile à l'allongement des délais de prescription. Aujourd'hui, ces dispositions font presque consensus, et je ne doute pas qu'il en sera de même, à l'avenir, pour la reconnaissance de l'incapacité absolue

de violences sexuelles commis sur mineurs qui nous aurait permis de sortir de la définition du viol. Je ne suis toujours pas convaincue que les mesures proposées dans ce texte sont de nature à protéger réellement les mineurs. C'est d'ailleurs ce qui conduira le groupe

à l'interruption de la prescription en cas de commission par leur auteur d'un même crime contre d'autres mineurs, la transformation du délit de non-dénonciation des mauvais traitements, des privations et des atteintes sexuelles commises à l'encontre de mineurs, ainsi que l'allongement du délai de prescription pour ce délit de six à dix ans. En ce qui concerne le renforcement de la protection des violences sexuelles sur mineurs, nous considérons que le texte modifié par notre Haute Assemblée comporte également quelques avancées. La vulnérabilité en ressort mieux définie, avec la prise en compte de la détresse économique et la création d'une circonstance aggravante d'ivresse stupéfiante. L'introduction de la possibilité pour les victimes de violences sexuelles de se faire accompagner d'un représentant d'une association conventionnée d'aide aux victimes dès le début du dépôt de la plainte est également une avancée importante. Enfin, le renforcement de la prévention grâce à une plus grande précision des textes relatifs aux obligations de signalement des médecins en cas de suspicion de violences psychologiques, physiques et sexuelles, répond aux préoccupations que nous avions évoquées lors de la discussion générale.

ayant pris part à ce débat qui, me semble-t-il, honore notre assemblée. Ce fut un débat approfondi. Nombre de points de vue convergents se sont exprimés ; certains points de vue divergents aussi, mais ils ont été généralement surmontés avec le meilleur état d'esprit, ce qui permet d'offrir à nos concitoyens l'image d'une assemblée délibérative qui va au fond des choses. Je voudrais

a permis à des représentants de tous les groupes politiques de se rassembler pour forger les positions de la commission des lois, exprimer de très larges consensus ; il avait déjà permis l'adoption par le Sénat

pour aller au-delà des frontières de chacun de nos groupes, ont été particulièrement dignes d'éloges, de même que sa sensibilité, qui doit sans doute beaucoup au métier qu'elle exerçait et continue partiellement à exercer, celui de médecin.

travail, et combien il a permis d'agréger encore, à partir de ce point de départ déjà marqué par beaucoup d'ouverture d'esprit, des points de vue jusqu'alors dissociés

tout, profondément et intimement. Nous avons fait de notre mieux. Cela ne suffira pas, mais nous avons au moins le mérite de porter sur la place publique l'horreur des violences sexuelles envers les mineurs, dont il faut oser parler et pour lesquels il faut briser le tabou. Nous comptons évidemment sur chacune et chacun d'entre nous pour porter ce combat.

Le scrutin est ouvert.